L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous venons tout juste d’achever l’examen du projet de loi d’orientation pour « grand » texte, au moins par sa taille, dont le parcours législatif a duré une année entière, nous nous penchons ce matin sur une proposition de loi le périmètre est beaucoup plus restreint et dont la gestation a été beaucoup plus rapide. Déposée fin novembre 2025 par la députée Nicole Le Peih, avec le concours du ministère de l’agriculture, elle a été examinée en commission mixte paritaire ce lundi ; nous devons maintenant en voter les conclusions. Cette « petite » proposition de loi relative au fonctionnement des chambres d’agriculture et de la Mutualité sociale agricole (MSA) n’en reste pas moins cruciale pour « l’exercice de la démocratie agricole », pour reprendre l’intitulé à répondre à une situation urgente : assurer la continuité du fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole et des chambres départementales d’agriculture, qui sont le cœur de notre démocratie agricole. Les bureaux des chambres d’agriculture doivent être constitués au plus tard le 5 mars. Or, en raison des incompatibilités prévues à l’article L. 254 1 2 du

dans les bureaux des chambres départementales d’agriculture et au conseil d’administration de la tête de réseau Chambres d’agriculture France. Premier concerné, son président Sébastien Windsor nous avait alertés de longue date sur cette problématique qui risquait de restreindre le vivier des professionnels éligibles. L’article 1 de la présente proposition de loi vise de remplacer une incompatibilité stricte par une règle de déport lors des délibérations relatives au conseil sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. C’était le cœur du texte. Il n’aura échappé à personne que les résultats de ces élections aux chambres d’agriculture, qui ont lieu tous les six ans, ont été proclamés en fin de semaine dernière. constate, cette fois ci, une stabilité de la participation – le niveau est exceptionnellement élevé pour des élections professionnelles –, mais aussi le basculement d’un certain nombre de chambres

agricole est bien vivante et que les listes minoritaires un jour peuvent devenir majoritaires un autre jour : eh oui, c’est aussi cela la démocratie Voilà pourquoi nous avons jugé inutile de maintenir dans le texte une demande de rapport, prévue par l’Assemblée nationale, sur l’opportunité d’introduire un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale pour les élections aux chambres d’agriculture, au moment même où ces élections se tenaient… Par ailleurs, en séance, un amendement de notre collègue Christian Redon Sarrazy a rétabli la condition, supprimée à l’Assemblée nationale, d’être à jour de cotisations pour être éligible comme délégué ou administrateur d’une caisse de MSA. Ce rétablissement a semblé véritablement tomber sous le sens. L’article 2 donne déjà aux agriculteurs en difficulté financière

C’est pourquoi je me félicite, monsieur le ministre, que la commission mixte paritaire, qui s’est réunie lundi à l’Assemblée nationale, ait entériné, à la quasi unanimité, le texte voté par le Sénat.

Pour conclure, il est clair que ce texte n’est qu’un premier pas. Je forme le vœu que les réformes plus substantielles proposées par le Sénat,

mesdames, messieurs les sénateurs, alors que les bureaux des chambres d’agriculture sont en voie de renouvellement à la suite des élections qui viennent de s’achever, la commission mixte paritaire est parvenue à trouver un accord sur la proposition de loi déposée par la députée Nicole Le Peih. C’est une excellente nouvelle pour nos élus agricoles Si elle est retenue par un impératif avec le Président de la République, Mme la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire tenait, monsieur le sénateur Louault, à vous remercier personnellement d’avoir conduit ces travaux à leur terme. Ce faisant, avec cette proposition de loi, nous acterons deux acquis démocratiques. Tout d’abord, vous permettez avec ce texte de ne plus exclure de la gouvernance des chambres les élus des coopératives.

Le second acquis concerne les élections à la Mutualité sociale agricole. La proposition de loi sur laquelle vous vous exprimerez prévoit de réarrimer les plus précaires à l’exercice de la démocratie sociale, en octroyant le droit de vote à ceux qui en étaient jusque là privés en raison du non paiement de leur cotisation depuis plus de six mois. Ce progrès démocratique trouvera à s’appliquer dès les élections de 2030. Mesdames, messieurs les sénateurs, grâce à votre texte, vous permettez de réadapter aussi les élections dans les chambres d’agriculture et à la MSA aux réalités territoriales. Je parle d’abord des dispositions permettant de sécuriser sur le plan administratif les élections à la MSA des délégués dans les ex cantons de la métropole de Lyon. Par ailleurs, et surtout, nous acterons le report d’un an des élections de la chambre d’agriculture de Mayotte. Le drame personnel et collectif que vivent les Mahorais ne nous permettait pas d’assurer la tenue des élections dans des conditions de sérénité suffisantes. Je compte donc sur votre responsabilité pour acter définitivement ce report. Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, en votant ce texte, nous actons des principes forts au cœur de la démocratie agricole. Je parle, bien sûr, des dispositions imposant la parité sur les listes pour les délégués cantonaux élus du deuxième collège du MSA de 2030 est un horizon ambitieux, compte tenu de l’inégale représentation des femmes et des hommes qui persiste aujourd’hui encore dans le secteur agricole, mais néanmoins réaliste. Votre texte apporte ainsi une pierre de plus à l’édifice de revalorisation de de la place et du statut des femmes en agriculture, un engagement très cher à Mme la ministre de l’agriculture. Mesdames, messieurs les sénateurs, en votant cette proposition de loi, nous offrirons à nos agriculteurs une respiration démocratique essentielle dans la période difficile qu’ils traversent sur le plan économique et social. Je vous appelle donc, bien entendu,

derniers. Lorsqu’il y a amalgame entre conseil et vente, le conseil peut vite devenir le moyen de doper la vente. La volonté du législateur était donc et demeure tout à fait louable. louable. Mais ce faisant, le législateur n’avait sûrement pas perçu que les diverses coopératives agricoles, créées par les agriculteurs eux mêmes pour défendre les productions à la ferme, et qui souvent vendent ces produits, seraient aussi concernées par cette disposition législative qui, de fait, allait empêcher ces agriculteurs de pouvoir être élus dans les organismes de direction d’un certain nombre d’institutions agricoles. Il convenait donc d’adapter la loi pour corriger cette injustice tout en assortissant cette adaptation d’un certain nombre de prescriptions ne remettant pas en cause les objectifs fixés par la loi Égalim de 2018.

Les élections dans les chambres d’agriculture viennent d’avoir lieu. Les désignations dans un certain nombre d’instances nationales devant intervenir dans les prochaines semaines, il était urgent de légiférer. C’est ce qu’il nous est proposé de faire aujourd’hui.

proposition de loi peu ambitieuse concernant le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la Mutualité sociale agricole. Comme je l’ai souligné la semaine dernière, ce texte ne constitue nullement une réforme en profondeur de la démocratie agricole, Il ne prévoit que des ajustements mineurs et n’aborde pas les véritables enjeux démocratiques qui s’imposent à nous. Je ne m’attarderai pas sur l’article 1, qui constitue pour nous un recul inacceptable. En remettant en cause la séparation entre la vente et le conseil en matière de produits phytosanitaires et en permettant aux élus des coopératives agricoles de siéger dans les instances dirigeantes des chambres d’agriculture, cette proposition de loi brouille dangereusement les lignes. Sous prétexte d’un manque de candidats dans certaines régions, elle tend à favoriser un mélange des genres préoccupant.

Il est donc impératif de repenser un système qui ne correspond plus aux attentes d’une partie significative de la profession, dont près de la moitié s’est abstenue lors des élections. Ce fonctionnement verrouillé empêche une prise en compte réelle des préoccupations de l’ensemble des acteurs du secteur, notamment celles des nouvelles générations d’agriculteurs, soucieuses de concilier production et respect de l’environnement.

Les résultats des récentes élections de janvier 2025 l’ont démontré : malgré un affaiblissement de la coalition FNSEA JA, le mode de scrutin lui permet de conserver 80 % des chambres en ayant recueilli moins de 50 % des suffrages. Plus grave, dans chaque chambre le pluralisme est quasi inexistant. Tant que ce système favorisera la majorité en place au détriment de l’expression d’autres sensibilités, malgré une diversité syndicale réelle, tant que le monde agricole ne pourra s’exprimer à travers un scrutin plus équitable, fondé sur la proportionnelle sans prime majoritaire excessive, le fonctionnement des chambres d’agriculture perdra en légitimité et en efficacité. Il était compréhensible de reporter ce débat en période électorale, mais désormais il ne peut plus être éludé. Les élections étant derrière nous, il est de notre responsabilité de repenser le cadre démocratique de nos chambres d’agriculture pour qu’il soit plus adapté aux défis actuels du secteur. Hier soir encore, les grandes orientations de notre agriculture pour la prochaine décennie ont été esquissées. Elles ne sont aucunement représentatives des attentes de la société, pas plus que de celles du monde agricole. D’autres sensibilités devraient pouvoir s’exprimer dans les chambres d’agriculture, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Il est désormais temps de réformer le mode de scrutin, de garantir un pluralisme effectif, de diversifier la composition des instances et d’assurer une répartition plus équitable des financements.

le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la Mutualité sociale agricole nous aura néanmoins permis de mettre fin à quelques dysfonctionnements et d’engager des débats importants.

acter le report des élections consulaires à Mayotte et à proroger le dispositif dérogatoire permettant le cumul au sein des chambres entre activités de conseil et activités de vente et de distribution de produits phytopharmaceutiques.

articles sur huit ayant été votés conformes au texte de l’Assemblée nationale, seuls deux articles restaient à discuter en notre amendement visant à réintroduire la condition d’être à jour depuis au moins six mois de ses cotisations sociales pour être candidat aux élections de la MSA a été adopté en séance et conservé dans le texte final. Il nous paraissait en effet nécessaire de rétablir cette disposition supprimée par l’Assemblée nationale. Si les considérations techniques ont été aisément réglées, c’est que les véritables points clivants n’ont trouvé aucune traduction législative dans ce texte.

Nous attendons donc les propositions du Gouvernement sur ce sujet pour freiner cette dérive monopolistique inquiétante, qui n’a rien de démocratique. Je reviendrai également sur la question de la séparation entre l’activité de vente et l’activité de conseil pour les produits phytopharmaceutiques, qui occupait l’essentiel de l’article 1. Nous n’avons formulé aucune opposition à la pérennisation du dispositif transitoire – le non cumul des deux fonctions n’ayant, de fait, jamais été appliqué en dépit de l’adoption de la loi Égalim. Néanmoins, nous avions souhaité l’assortir de quelques garde fous qui auraient permis de renforcer l’application de la règle du déport, indispensable pour autoriser ce cumul. À ce jour, il n’existe en effet aucune sanction en cas de non respect de cette obligation, ce qui est pour le moins surprenant et laisse libre cours à de potentielles dérives. Notre amendement visant à prévoir une contravention n’a pas été adopté, et nous le regrettons. Faut il revoir totalement le système ? La question a été posée par les députés socialistes. Le débat reste donc ouvert, tout comme celui sur la représentativité des agriculteurs au sein des instances agricoles,

être pas la politique agricole française, comme une grande loi d’avenir ou d’orientation. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle était utile et urgente. Elle a le mérite, une fois n’est pas coutume, de mettre tout le monde d’accord. Comme nous l’avons souligné à de multiples reprises, ce texte est essentiellement technique. Circonscrit au nécessaire, il permettra le bon déroulé des élections actuelles et à venir dans les chambres d’agriculture,

L’Assemblée nationale a adopté ce texte hier. Nous allons à présent l’adopter à notre tour. Dès lors, certaines adaptations pourraient entrer en vigueur avant la date butoir pour l’installation des nouveaux bureaux des chambres d’agriculture. notamment à l’article 1, qui vise à permettre aux associés coopérateurs et aux membres de coopératives vendant des produits phytopharmaceutiques de participer aux instances dirigeantes des chambres d’agriculture. Il est en effet absurde, d’un côté, de vouloir les exclure des instances dirigeantes et, de l’autre, de demander un fonctionnement plus démocratique aux chambres ! Cette rectification était nécessaire et urgente au vu du calendrier.

pour autant un retour en arrière. Ce n’est pas souhaitable ! Pour autant, il est impératif de retravailler ce mécanisme dans un futur texte. Encore une fois, ce n’est pas l’objet de cette proposition de loi. Je tiens, au passage, à saluer les agriculteurs qui se sont présentés aux élections et qui ont été élus. Je les remercie pour leur engagement en faveur du monde agricole. Les résultats sont contrastés et témoignent de la colère de certains.

de loi permettra demain aux agriculteurs vendant des produits phytopharmaceutiques d’être également élus au bureau des chambres d’agriculture. Le texte vise à instaurer, en parallèle, une règle de déport lorsque les chambres procèdent à des travaux et délibérations concernant l’activité de conseil sur l’utilisation de ces produits. Cette évolution est une réelle avancée. Elle revient sur une incohérence de la loi Égalim.

Cette mesure est cruciale pour enfin traiter les agriculteurs comme tous les autres acteurs économiques. Nous légiférons ce matin avec la conscience de l’urgence que commande la situation urgence de la procédure, qui a conduit le Parlement à adopter cette proposition de loi en un temps record, avant le renouvellement du bureau des chambres d’agriculture ; urgence des attentes exprimées par les agriculteurs depuis plus d’un an, exaspérés par une réglementation qui désespère et qui contraint plus qu’elle ne libère ; urgence des réponses attendues de la part des pouvoirs publics, alors qu’un vote clairement contestataire s’est exprimé dans les urnes lors du renouvellement des chambres d’agriculture

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons plus traiter l’agriculture avec cette forme de paternalisme condescendant que l’on a trop souvent entendue lors des récents L’agriculture ne peut plus être traitée à l’aune de son poids dans notre PIB. Elle conditionne notre indépendance et notre souveraineté alimentaire à l’avenir. Elle est l’un des meilleurs remèdes aux problèmes de compétitivité de notre pays et l’assurance de notre biodiversité et de nos paysages. N’oublions pas non plus que l’agriculture est un tissu économique vital pour l’équilibre et le développement de nos territoires. La France ne pourra pas tenir dans la compétition mondiale avec une économie uniquement fondée sur les services Le retour de la puissance française passe par la restauration de notre puissance agricole. Bravo ! Tout à fait ! Les membres du groupe Les Républicains voteront bien entendu le texte issu de l’accord en CMP. Ils veulent redire leur attachement à cette forme originale de démocratie agricole que sont les chambres d’agriculture

de notre collègue députée Nicole Le Peih. Ce texte, au delà de ses aspects techniques, répond à des enjeux fondamentaux pour l’avenir de notre agriculture et, plus particulièrement, pour le fonctionnement de nos chambres d’agriculture. Ces dernières jouent un rôle clé dans l’organisation et l’évolution du monde agricole. Elles constituent un véritable trait d’union entre l’État et les agriculteurs. offrent un accompagnement essentiel, un cadre de dialogue structurant et sont une force de proposition pour l’avenir de notre modèle agricole. Elles rassemblent l’ensemble des acteurs du secteur : exploitants, propriétaires, salariés, organisations professionnelles, coopératives, syndicats et organismes spécialisés. les chambres d’agriculture puissent fonctionner de manière efficiente et adaptée aux défis actuels. Or nous constatons que certaines dispositions réglementaires ne correspondent plus aux réalités du terrain. Cette proposition de loi vise donc à moderniser et à clarifier leur gouvernance pour la rendre plus efficace, plus transparente et plus en phase avec les évolutions du secteur. Tout d’abord, ce texte corrige une incohérence issue de la séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytosanitaires. Jusqu’à présent, la réglementation empêchait les administrateurs de coopératives agricoles de siéger au sein des bureaux des chambres d’agriculture, situation paradoxale qui privait ces instances de l’expertise et de la connaissance précieuse de ces acteurs majeurs du monde agricole. En rétablissant la possibilité pour eux d’y siéger, nous garantissons une gouvernance plus équilibrée et représentative de la diversité du secteur. Ensuite, ce texte introduit une disposition de bon sens, en rendant obligatoire l’adoption d’un règlement intérieur dans chaque chambre d’agriculture. Il s’agit d’un élément fondamental pour assurer une gestion transparente et démocratique du fonctionnement interne des chambres. Ce cadre garantira une plus grande stabilité et une meilleure lisibilité des pratiques au sein de ces institutions. Par ailleurs, la proposition de loi s’inscrit dans l’effort constant de simplification que le Sénat défend. Elle facilite notamment la participation des exploitants agricoles aux élections des délégués et des administrateurs de la Mutualité sociale agricole. Aujourd’hui, les agriculteurs débiteurs de cotisations depuis plus de six mois sont exclus du processus électoral, ce qui pose de nombreuses difficultés pratiques et juridiques : cela complique : cela complique la constitution des listes électorales de la MSA, en excluant des exploitants parfois pour de simples raisons administratives. En levant cette restriction, nous garantissons une participation plus large et plus juste des agriculteurs à la gouvernance de leur système de protection sociale. Par ailleurs, ce texte sécurise l’organisation des élections des membres de la MSA pour 2025, en harmonisant les dates des différents scrutins, ce qui constitue une avancée bienvenue pour la lisibilité et l’organisation de ces échéances importantes. Enfin, le groupe RDPI se félicite que la commission mixte paritaire ait décidé de maintenir la suppression de l’article 1,

Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale voilà quelques jours, ce texte est essentiellement technique. Il s’attache seulement à faciliter le déroulement des élections au sein des chambres d’agriculture et de la Mutualité sociale agricole, en apportant des solutions pragmatiques et logiques aux problèmes qu’elles soulèvent.

Pourtant, les enjeux de pluralisme et de représentativité, qui ne sont pas évoqués ici, ont eu un écho important lors des élections au sein des chambres d’agriculture.

Nous ne pouvons nier la réalité du terrain : trop d’exploitants se sentent oubliés et sous représentés. Faut il rappeler le taux de participation à ces élections pour s’en convaincre ? Il y a six ans, moins d’un agriculteur sur deux avait voté,

les 2,2 millions d’électeurs, dont près de 400 000 chefs d’exploitation, mais aussi des retraités, des salariés ou des propriétaires fonciers, étaient appelés à élire leurs représentants par voie électronique ou postale. Le monde agricole a besoin de changement, et celui ci doit passer par plus de transparence et de reconnaissance. La confiance dans les partis politiques comme dans les syndicats continue de reculer,

La Cour des comptes a d’ailleurs appelé, dans son rapport public de 2021, à une refonte du mode d’élection pour favoriser la pluralité syndicale. Dans un rapport

sociale méritée. Le décalage est criant entre la vocation de l’agriculteur – nourrir la population – et sa juste reconnaissance tant économique que sociale ou politique. politique. Ce texte permet au moins de maintenir la règle du déport, rendue obligatoire depuis le 1 janvier 2021 dans les chambres d’agriculture et indispensable pour préserver les objectifs de prévention et de lutte contre les conflits d’intérêts. Surtout, ce texte rétablit une égalité de traitement entre les agriculteurs en ouvrant le droit de candidater et de voter à tous les adhérents à la MSA en âge de voter, même s’ils ne sont pas à jour de leurs cotisations sociales. Cette limitation du droit de vote, en plus de ne pas être évidente ni conforme au principe d’égalité devant la loi, ainsi qu’à la règle de l’égalité du suffrage énoncée à l’article 3 de la Constitution, constituait une double peine pour des agriculteurs déjà confrontés à des difficultés sociales et économiques importantes.

projet de loi d’orientation agricole… Sans oublier les discussions à venir sur un futur texte Égalim ! La présente proposition de loi est le dernier texte de cette intense séquence. Rarement les questions agricoles ont été à ce point au premier plan de l’agenda législatif, et pour cause notre souveraineté alimentaire est en danger et nous devions évidemment faire de cette question une priorité nationale. Au sortir des élections des chambres d’agriculture et à quelques jours de l’ouverture du Salon de l’agriculture comme des élections à la MSA, ce texte technique est important pour le nouveau cycle de démocratie agricole qui s’ouvre en 2025, dans un climat de contestations majeures. l’exercice du métier d’agriculteur dans « l’après » conseil stratégique en agriculture, actant les aménagements à la séparation entre les activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques.

À quelques semaines de la constitution des bureaux des chambres d’agriculture, ce texte arrive juste à temps et nous permettra de continuer à bénéficier de l’expertise de personnes ancrées dans l’écosystème dont s’est dotée notre agriculture depuis de nombreuses années. fois les urgences techniques traitées, il faut revenir à des débats politiques au long cours sur le rôle des chambres d’agriculture. Je pense aux débats que nous avons eus sur le rôle et le périmètre du guichet France Services Agriculture, notamment ces derniers jours, mais également sur l’après conseil lors de nos discussions sur la proposition

reçoivent des injonctions contradictoires, qui deviennent inaudibles. Mes chers collègues, nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité. J’en veux pour preuve les trop longs débats que nous avons eus, ces derniers jours, sur la hauteur, la largeur et la taille de la haie ou encore sur le bien être des chiens des chiens de troupeaux. Il y a parfois de quoi se décourager, mais je veux rester optimiste. Il me semble que nous devrions prendre un peu de recul et nous montrer à la hauteur du défi que nous avons à relever et des attentes de nos agriculteurs, qui comptent encore sur nous.

deux mois après le cyclone Chido, j’exprime de nouveau à mes compatriotes mahorais toute ma sympathie et toute ma solidarité dans l’épreuve qu’ils traversent. Pour eux, nous avions à cœur de faire aboutir le projet de loi d’urgence pour Mayotte et de nous atteler rapidement à la reconstruction C’est cet esprit de responsabilité qui a présidé aux travaux de la commission mixte paritaire. Avec Isabelle Florennes, rapporteure pour avis de la commission des lois, et Christine Bonfanti Dossat, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, nous avons travaillé de concert au compromis trouvé lundi dernier, qui préserve la grande majorité des apports du Sénat. Nous pouvons nous en féliciter. En tant que chambre des territoires, nous avons eu pour boussole l’association étroite des élus mahorais à la reconstruction. je salue mes collègues sénateurs de Mayotte, Salama Ramia et Saïd Omar Oili. Je me réjouis que les acquis du Sénat s’agissant de la représentation des collectivités dans la gouvernance de l’établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte Pour que la reconstruction soit acceptée de tous, il est essentiel d’assurer la coopération entre l’État, principal financeur, et les acteurs locaux. Je les ai tous rencontrés lors de mon déplacement à Mayotte à la fin du mois de janvier : ce sont eux qui détiennent les clés de la compréhension de leur territoire et de ses contraintes. La reconstruction doit être accompagnée d’un effort résolu contre le retour des bidonvilles. C’est pourquoi la CMP a maintenu l’encadrement de la vente de tôles, ainsi que l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter les règles de lutte contre l’habitat illégal.

ciblé sur le logement temporaire des personnes venues en renfort, les bureaux et les salles de classe temporaires. Ces constructions ne pourront pas être implantées sans l’accord du maire. La CMP a entériné cette solution équilibrée et sécurisée. Au delà des bidonvilles, il nous fallait tenir compte du fait que deux tiers des constructions à Mayotte ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme. Retenant là encore un acquis du Sénat, la CMP a étendu le droit à la reconstruction à l’identique à l’ensemble des bâtiments en dur datant d’avant 2013. Enfin, afin de soutenir financièrement les ménages et les entreprises, les dispositifs introduits au cours de l’examen du texte au Sénat, comme le prêt à taux zéro pour la reconstruction des logements ainsi que l’exonération de taxe générale sur les activités En guise de compromis entre les deux chambres, le plafond de la réduction d’impôt pour les dons en faveur des victimes a quant à lui été ramené à 2 000 euros. Bien sûr, ce texte n’a pas la prétention de répondre à toutes les difficultés des Mahorais. Ces difficultés, nous les connaissons un niveau de pauvreté inégalé, la prolifération de l’habitat informel, une insécurité alimentée par une immigration clandestine massive. Je crois donc essentiel de nous préparer d’ores et déjà à la prochaine étape : le projet de loi de programmation pour Mayotte annoncé par le ministre d’État, ministre des outre mer.

mais il est indispensable pour poser les bases d’une reconstruction à la fois rapide, pérenne et concertée. Telles sont, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’urgence pour Mayotte. J’espère que vous les approuverez très largement. Bravo ! La parole

l’absence aujourd’hui de M. le ministre d’État, ministre des outre mer, Manuel Valls, retenu actuellement auprès du Président de la République pour une réunion sur la Nouvelle Calédonie. Il y a quelques semaines, lorsqu’il présentait ce projet de loi d’urgence pour Mayotte devant la commission des affaires économiques de votre assemblée, il avait souhaité, plus largement, définir la méthode du Gouvernement, laquelle s’organise en trois temps : les urgences vitales, la reconstruction, la refondation. Sur le premier temps – la gestion de crise –, nous pouvons dire, avec lucidité, que nous nous dirigeons progressivement vers une sortie de la phase d’urgence vitale. Des difficultés persistent, mais l’accès à l’électricité ou à la nourriture s’est vraiment amélioré. L’objectif de rétablissement de l’électricité à 100 % au 31 janvier a été tenu. La rentrée scolaire s’est faite, dans des conditions difficiles certes, mais l’engagement des personnels éducatifs et des renforts de sécurité civile a permis de l’organiser. Dans le second degré, l’intégralité des établissements a rouvert. Dans le premier degré, seule une vingtaine d’écoles demeurent dans l’incapacité d’accueillir les élèves, des « tentes écoles » ont été positionnées. En outre, 1 100 élèves ont pu être scolarisés hors de Mayotte, dont 400 à La Réunion. Par ailleurs, vous le savez, nous aménageons les épreuves de fin d’année et les remplaçons en grande partie par du contrôle continu. La reconstruction des écoles est une priorité. C’est pourquoi le projet de loi de finances pour 2025 prévoit 2,5 millions d’euros mobilisables immédiatement.

Ces avancées sont évidemment dues aux agents de l’État et, en premier lieu, au préfet François Xavier Bieuville, aux volontaires et aux bénévoles mobilisés, mais, surtout, à l’engagement des Mahorais : la population, bien sûr, mais aussi les entrepreneurs, que l’État accompagne sans réserve. La circulaire sur le fonds de secours outre mer, qui prévoit notamment 15 millions d’euros d’aides pour les agriculteurs, a été signée par l’ensemble des ministres concernés. Je tiens aussi à rendre hommage aux élus. Impliqués dans la gestion de la crise, ils seront incontournables dans la reconstruction et la refondation qui nous attendent. C’est pourquoi le ministre d’État a signé, lors de son dernier déplacement à Mayotte, avec le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni, et le président de l’association des maires de Mayotte, Madi Souf, une convention d’intention affirmant les grands principes devant guider la refondation durcissement des règles contre l’immigration illégale, lutte contre les bidonvilles, développement des infrastructures, convergence économique et sociale. Nous nous éloignons donc progressivement Pour autant, tout reste à faire ! La gestion de crise passée, il nous faut reconstruire, puis refonder Mayotte. De nombreux défis sont devant nous. Sur la reconstruction – le deuxième temps que j’évoquais au début de mon propos –, nous franchissons aujourd’hui une étape décisive. Face au chaos, nous avions collectivement, dans le cadre de ce projet de loi, une responsabilité extrêmement forte. Le Parlement s’est hissé à la hauteur de cette responsabilité. D’abord, ce projet de loi a été adopté en première lecture à la quasi unanimité de l’Assemblée nationale et à l’unanimité du Sénat. Ensuite, la commission mixte paritaire n’a eu aucun mal à trouver un accord utile et équilibré, et nous en remercions très sincèrement ses deux rapporteurs. Sur le fond, des compromis féconds ont été trouvés par les deux chambres. trouvés par les deux chambres. Ainsi, à l’article 1, la composition de l’établissement public de reconstruction a d’ores et déjà été précisée afin d’assurer une meilleure représentation des collectivités territoriales, notamment des intercommunalités ; à l’article 2, la prise en charge par l’État de la reconstruction des écoles se fera à la demande des communes concernées enfin, la dispense de toute formalité d’urbanisme pour les constructions démontables temporaires de l’article 3 a été davantage encadrée afin de limiter leurs utilisations possibles et de garantir clairement qu’elles ne deviendront pas pérennes. Outre ces modifications des articles initiaux, des mesures ont également été ajoutées au cours du débat parlementaire, sur des sujets fondamentaux pour nous. Plusieurs dispositifs de lutte contre les bidonvilles ont été intégrés, sur l’initiative ou avec le soutien du Gouvernement, comme l’extension du champ de l’ordonnance de l’article 4 ou ou l’encadrement de la vente de tôles aux particuliers à l’article 4. L’article 13 AA permettra de garantir la participation des entreprises mahoraises à la reconstruction, puisqu’il prévoit la faculté de réserver jusqu’à 30 % du montant estimé d’un marché aux microentreprises, PME et artisans basés à Mayotte. L’article 17 AA, intégré au texte sur l’initiative du Gouvernement, met en place un prêt à taux zéro ouvert à toutes les familles mahoraises pour reconstruire leur maison, même lorsque leur habitation n’était pas assurée. Il permettra d’emprunter jusqu’à 50 000 euros, pour une durée maximale pouvant atteindre trente ans, avec un différé d’amortissement de cinq ans. Le Gouvernement s’engage à ce que ce prêt soit distribué le plus rapidement possible, avec les banques et Action Logement. Enfin, l’article 17 exonère le territoire de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets pendant deux ans. Tous ces ajouts témoignent de la richesse du débat parlementaire. La reconstruction nécessitera des engagements financiers considérables. La mission interinspections chargée d’évaluer les dégâts achève ses travaux. Le coût des destructions se situera entre 3 et 3,5 milliards d’euros. L’État sera au rendez vous, en octroyant des aides directes et en mobilisant des fonds européens, et ce sur plusieurs années. Les assurances et l’Agence française de développement auront aussi un rôle à jouer. Et je l’ai dit, ce projet de loi garantit aussi la participation des entreprises mahoraises à la reconstruction de leur territoire. Le Gouvernement tout entier est mobilisé pour faciliter cette reconstruction. Le ministre d’État Manuel Valls et le ministre des armées, Sébastien Lecornu, ont décidé de créer un bataillon temporaire de reconstruction, doté de plusieurs compagnies de génie, d’infanterie, de commandement et de logistique. Ce sont entre 350 et 400 soldats qui iront ainsi s’installer à Mayotte. Ce projet de loi, que vous vous apprêtez à adopter définitivement, n’est qu’une première réponse, car, après le temps de l’urgence et celui de la reconstruction, viendra celui de la refondation. D’ici à quelques semaines, le ministre d’État, ministre des outre mer, présentera un second texte : un projet de loi de programmation pour Mayotte visant à permettre le développement économique, éducatif et social du territoire sur de nouvelles bases. Il s’appuiera sur le plan stratégique que va élaborer le général Facon, préfigurateur de l’établissement public et, surtout, chef de la mission interministérielle de reconstruction de Mayotte installée auprès du ministre d’État. Celui ci est de nouveau sur place, avec une partie de son équipe. Le Gouvernement sera notamment particulièrement attentif à ce que nous portions un véritable projet d’avenir, dirigé vers la jeunesse. Le régiment du service militaire adapté (RSMA) effectue déjà un travail remarquable. Des jeunes sont d’ores et déjà formés, dans ce cadre, aux métiers du raccordement à la fibre, par exemple. Si le cyclone a ravagé Mayotte, il a surtout révélé et exacerbé des calamités qui existaient déjà : un sous développement des infrastructures économiques et des services publics, entretenu par deux fléaux qui rongent l’île depuis des années : l’habitat illégal et l’immigration clandestine. de l’eau, par exemple, à défaut de changement structurel, nous reviendrons, au mieux, à la situation très insatisfaisante de l’avant Chido. C’est pourquoi, parmi les priorités du plan Mayotte debout figurent la construction d’une deuxième usine de dessalement et l’accélération de la création d’une troisième retenue collinaire. Nous avançons sur ces deux projets. Nous devons être très attentifs, car le risque d’une nouvelle crise de l’eau, semblable à celle de 2023, existe bel et bien. En matière de reconstruction de logements, d’infrastructures, d’entreprises ou de services publics, la zone franche globale sera Cependant, les maires et les entrepreneurs le disent tous : leurs projets sont empêchés par les bidonvilles. Soyons clairs : le Gouvernement ne laissera pas Mayotte redevenir une île bidonville.

Il faut aussi s’attaquer très sérieusement à l’immigration illégale, qui pèse sur tous les aspects de la vie quotidienne de nos compatriotes, nourrit l’ultraviolence et alimente des réseaux de trafiquants d’êtres humains.

l’allongement de la durée de résidence régulière des parents pour permettre l’accès des enfants à la nationalité française, l’amélioration des outils pour lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité ou l’encore l’extension de l’aide au retour volontaire des ressortissants africains dans leur pays d’origine. Nous devons porter le nombre d’éloignements de clandestins de 25 000 aujourd’hui à 35 000 demain. Cela suppose un rapport très ferme avec les autorités

Vous prouverez aux Mahorais que nous ne transigerons sur rien pour reconstruire l’île sur des bases plus saines, pour changer son visage et, à travers elle, leur vie tout entière. Nous passons commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire,

un peu plus d’une semaine, le Sénat adoptait à l’unanimité le projet de loi d’urgence pour Mayotte. Je ne reviendrai pas en détail sur les dispositions prévues dans le texte. Celui ci prévoit un certain nombre d’assouplissements et de dérogations, en matière, par exemple, de commande publique, avec un unique objectif

Ce texte, nous le savons tous, ne permettra pas de résoudre l’ensemble des problématiques de l’archipel. Son ambition est plus modeste : il s’agit uniquement de répondre aux dégâts immédiats provoqués par le passage du cyclone.

tant les enjeux sont grands et tant l’attente de la population se fait vive. Nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner le texte de compromis résultant des travaux de la commission mixte paritaire. Je considère qu’il est satisfaisant et qu’il conserve une grande partie des apports du Sénat,

demande des communes. Cet apport de la Haute Assemblée garantira sans aucun doute le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce dispositif a été complété a été complété en commission mixte paritaire, toujours dans l’optique de mieux assurer le respect des libertés locales, afin d’imposer le recueil de l’avis conforme des communes avant la construction de nouvelles écoles ou l’ouverture de nouvelles classes, ce dont je me satisfais également. également. Sur les articles relatifs à la commande publique, je tiens d’abord à souligner le maintien dans un article unique, introduit sur l’initiative du Sénat, de l’ensemble des des dispositions visant à favoriser les petites entreprises mahoraises lors de l’attribution des marchés publics destinés à reconstruire Mayotte. Ces dispositions seront sans aucun doute source de clarté pour les acteurs locaux. Je me réjouis par ailleurs du non rétablissement des mesures visant à limiter le recours à la sous traitance dans le cadre des marchés publics conclus pour reconstruire l’archipel, qui avaient été supprimées par le Sénat. Ces dispositions auraient en pour effet de pénaliser les petites entreprises mahoraises, voire de les évincer des marchés publics. Ces sociétés ont en effet souvent accès à la commande publique par le biais de la sous traitance.

Malheureusement, deux mois après le cyclone Chido, à Mayotte, et dix mois après les émeutes en Nouvelle Calédonie, la solidarité peine à se manifester et l’urgence est toujours d’actualité.

ayant fait preuve de solidarité envers les Mahorais sinistrés. Nous exprimons toutes nos condoléances aux proches des victimes et notre soutien aux personnes touchées, ainsi qu’à tous ceux qui leur portent secours. Mes chers collègues, alors que nous nous apprêtons à voter un projet de loi pour la reconstruction de Mayotte, nous le savons, il faudra faire beaucoup mieux qu’avant Chido. Il ne suffira pas de mener des opérations de destruction et d’expulsion massive des bidonvilles, comme a pu le faire l’ancien ministre de l’intérieur

de construire plusieurs centaines de milliers de logements pour les Mahorais qui peuplent ces bidonvilles. Il y va de la dignité et de la vie de ces personnes, qu’elles possèdent ou non des papiers. Ou la dignité humaine vaut pour tout le monde, ou elle ne vaut pour personne. Rappelons le, à Mayotte, avant le cyclone, plus du tiers des logements étaient des habitats de fortune, majoritairement en tôle.

qui ont cours uniquement sur des demi journées, par rotation. Les conséquences sur l’éducation d’une population âgée de moins de 20 ans à plus de 55 % sont graves. C’est pourtant là que se prépare l’avenir de l’île. Aussi, mes chers collègues, il revient au Sénat de ne pas tomber dans le piège de la division et de garantir à chacun En tant que Kanak, je connais trop bien cette facilité que sont le mépris et l’ignorance depuis l’Hexagone. Mon peuple en a payé un lourd tribut. Ce drame horrible nous permet de reconstruire Mayotte sur des bases solides et plus égalitaires. Ne souillons pas cet espoir par de la xénophobie stérile. Soyons à la hauteur des enjeux de l’Histoire.

Vous êtes chez vous, la nuit, à la campagne. À quelques kilomètres de là éclate un cataclysme naturel, une catastrophe naturelle, soit l’incendie, soit l’inondation. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants sont là qui fuient à travers champs, demi nus, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. « Votre maison est peut être déjà pleine, c’est possible, mais quand ils frappent à votre porte, vous la leur ouvrez et vous ne leur demandez pour ni leurs pièces d’état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccins. « Il y a là un devoir d’humanité élémentaire, je dirais presque, si les mots n’avaient pas l’air de jurer ensemble, ensemble, d’humanité animale. « Naturellement, ces malheureux ne pourront pas rester toujours là, c’est entendu. « Naturellement, il faudra trouver des solutions ayant un caractère de stabilité et de durée, mais enfin pour l’instant, en attendant qu’eux mêmes ailleurs trouvent un gîte plus sûr et plus durable, comment allez vous leur refuser l’asile d’une nuit ? » Ces mots ne sont pas de moi. Ils ont été prononcés

Je veux insister sur l’article 4 . Nous en avons longuement parlé dans cet hémicycle. Comment accepter de voter un texte qui conditionne l’achat de matériaux de construction, même s’il s’agit de tôles, à la présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ? Les registres d’identité et d’adresse ne font pas partie de notre identité écologiste. L’obligation de justifier d’une adresse pour construire ou reconstruire son habitat après un cyclone ne correspond ni à notre vision de l’égalité ni à notre conception de l’humanisme. Notre humanisme s’exprime également par la manière dont nous traitons nos enfants. À Mayotte, plus de la moitié des élèves suivent un enseignement en rotation et seulement deux jours par semaine.

Notre humanisme s’exprime aussi au travers de la protection du vivant et de notre biodiversité. Les outre mer représentent 80 % de la biodiversité française. L’archipel de Mayotte est un patrimoine naturel d’exception, terrestre comme marin

sans anticiper les aléas climatiques futurs ni intégrer un nouveau paradigme en matière d’impact énergétique et climatique. Alors nous nous sommes beaucoup questionnés. Allons nous voter ce texte si imparfait, nous qui refusons profondément de cautionner un projet qui manque de cœur, d’humanité et de vision durable ?

Cependant, nous avons bien pris note de l’engagement du Gouvernement de mettre en œuvre une véritable concertation avec les élus sur le contenu de cette ordonnance stratégique pour la suite du redressement de notre archipel.

sur les textes qui définiront en grande partie les conditions de la gouvernance de la reconstruction de ce territoire meurtri par le cyclone Chido et la tempête tropicale Dikeledi.

tout notre archipel, et le sentiment d’abandon est très largement répandu chez les Mahoraises et Mahorais. Afin d’éviter que le fossé entre l’Hexagone et notre archipel ne s’agrandisse, il faut impérativement que l’État tienne ses promesses.

La semaine dernière, j’ai assisté au départ d’un conteneur de la ville de Saint Denis pour Mayotte. L’ONG humanitaire Outre mer solidarités catastrophes avait collecté des tonnes de produits essentiels pour la population mahoraise.

en urgence, se concrétisent sur le terrain. Nous resterons fidèles à la devise que tous les Mahorais connaissent et qui constitue un emblème de notre relation avec les autorités nationales :, en shimaoré

par une loi soutenue par Joseph Faure, premier sénateur paysan. Il était corrézien ! Il y a trois jours, la CMP sur le projet de loi d’urgence pour Mayotte parvenait à un accord.

Nous parlons en effet de l’une des catastrophes naturelles les plus graves qu’a connues notre pays depuis près d’un siècle. On plus de 4 000 blessés. Les maisons de centaines de milliers de personnes ont été détruites, les entreprises et l’agriculture ravagées, l’hôpital, l’aéroport, les routes, la préfecture ou encore les établissements scolaires De nouveau, nous tenons à adresser toutes nos pensées aux victimes du cyclone et à leurs familles. Reconstruire, vite et bien, c’est la priorité pour le territoire mahorais, qui doit se relever. a déjà commencé à faire face à ce défi avec résilience et nous devons continuer de l’accompagner au mieux. c’est tout l’objet de ce texte, qui instaure de nombreuses dérogations au droit commun en matière d’urbanisme. Elles permettront, notamment, de simplifier les procédures, de raccourcir certains délais et d’assouplir les règles des marchés publics. C’est indispensable pour avancer.

de loi assure ainsi la représentation des maires dans le conseil d’administration du nouvel établissement public chargé de la coordination des travaux de reconstruction. Comme vous, madame le rapporteur, rapporteur, nous pensons que la réussite de la reconstruction passera par l’association étroite des élus locaux. Les propriétaires pourront en outre bénéficier d’un prêt à taux zéro pour réhabiliter leur logement, dans la limite de 50 000 euros.

Plusieurs mesures permettront en effet à de nombreuses personnes de bénéficier, temporairement, du renouvellement automatique de certaines prestations sociales et des allocations des allocations chômage jusqu’au 30 juin 2025. De plus, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues depuis le passage du cyclone par les entreprises et les travailleurs indépendants sera temporairement suspendu. Nous avons eu l’occasion de le dire, ce projet de loi est un texte d’urgence qui n’a pas vocation à régler les problèmes structurels de Mayotte, lesquels sont largement antérieurs au passage du cyclone. Ces difficultés sont aussi nombreuses d’accès à l’eau et aux soins, chômage, pauvreté, immigration illégale massive… Prouvons aux Mahorais que nous les avons entendus et que nous allons enfin agir sur ces sujets qui rongent le territoire depuis trop longtemps. J’entends souvent rappeler, à juste titre, que les outre mer, c’est la France. Mayotte, c’est la France. Mais cette année, monsieur le ministre, mes chers collègues, au delà des mots, il nous faudra agir, et vite, pour le prouver. Notre groupe votera évidemment ce texte. La parole est

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, deux mois après le cataclysme qui a frappé Mayotte, nous arrivons aujourd’hui au terme de l’examen parlementaire de ce texte d’urgence et de reconstruction. Élaboré en quelques jours, puis présenté par le Gouvernement début janvier, ce projet de loi a été transmis le 22 janvier au Sénat, où nous avons tous eu à cœur de le faire aboutir le plus rapidement possible. Nous le devions à nos compatriotes mahorais. Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire réunie lundi dernier sur le texte soit parvenue à un accord. Je tiens très sincèrement à remercier les rapporteurs, Micheline Jacques, rapporteur au fond de la commission des affaires économiques, Christine Bonfanti Dossat, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, et Isabelle Florennes, rapporteure pour avis de la commission des lois, qui ont effectué un travail essentiel sur un texte technique, dans des délais très courts. Le compromis auquel elles sont parvenues avec l’Assemblée nationale préserve la plupart des acquis du Sénat, notamment l’association des acteurs locaux, chère à notre assemblée. à ce sujet, à souligner le travail accompli par Micheline Jacques, qui s’est rendue sur place, à Mayotte. Son expérience de terrain a été précieuse pour enrichir le texte, de même que celle de nos collègues sénateurs de Mayotte, que je salue, Salama Ramia et Saïd Omar Oili, dont je connais l’engagement pour ce territoire. Le Sénat a eu à cœur d’aller au delà de la reprise des mesures

en matière d’urbanisme et de construction. Je rappelle en effet que deux tiers des constructions y ont été réalisés sans autorisation et que les habitations de fortune y représentent près d’un tiers du parc de logements. C’est également la raison pour laquelle nous saluons le fait que ce texte inclue dans le champ de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances des mesures pour favoriser la lutte contre l’habitat illégal à Mayotte, celui ci étant, nous le savons tous, un véritable fléau. Face à un cyclone qui a dévasté les logements, les outils de production, les infrastructures et les services publics, le contexte économique particulièrement dégradé a justifié l’adoption de mesures de soutien financier aux ménages et aux entreprises. Le Gouvernement a notamment instauré un prêt à taux zéro pour la reconstruction et la réhabilitation des logements, que nous avons naturellement conservé. En prenant en compte les spécificités du territoire mahorais, nous sommes parvenus à un texte opérationnel qui porte des mesures concrètes et adaptées aux réalités du terrain. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il faut maintenant entrer dans le temps long de la reconstruction. À cet égard, je salue l’annonce par M. le ministre d’État d’un projet de loi de programmation pour Mayotte dans les prochaines semaines. Au delà du cyclone Chido, qui les a mis rudement à l’épreuve, les Mahorais font face à des difficultés structurelles que nous connaissons bien, au premier rang desquelles figure l’insécurité. Le volet institutionnel et régalien de ce projet de loi de programmation sera sans doute essentiel. Pour autant, monsieur le ministre, je vous invite à ne pas négliger le volet économique. Des mesures pérennes et structurantes d’adaptation sont très attendues par les acteurs économiques locaux. Je pense notamment à la prise en compte des contraintes de l’insularité pour le développement de l’offre de logements abordables à Mayotte, structurellement insuffisante, ainsi qu’aux nécessaires mesures de soutien au tissu industriel et agricole local afin de favoriser le développement économique de l’archipel. Une délégation de la commission des affaires économiques se rendra à Mayotte à la fin du mois de mars. Ce déplacement est à notre sens essentiel essentiel pour préparer l’examen de ce texte au plus près du territoire, en concertation, bien sûr et toujours, avec les acteurs locaux. Mes chers collègues, en attendant ce second temps parlementaire, l’approbation large et sans ambiguïté de ce projet de loi d’urgence est nécessaire pour apporter le plus rapidement possible de premières réponses concrètes aux Mahorais. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains approuvera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’urgence pour Mayotte. Bravo ! La parole

dans ce département français de l’océan Indien. Ce drame humain et matériel a mis à l’épreuve notre capacité collective à répondre sans délai à l’urgence et à poser les bases d’une reconstruction durable de Mayotte. Face à l’ampleur de la catastrophe, il était de notre responsabilité de doter Mayotte d’un cadre législatif adapté à une reconstruction à la fois efficace et pérenne, respectueuse des réalités locales, des attentes des élus et de nos compatriotes mahorais. C’est dans cet esprit que députés et sénateurs ont travaillé au sein de cette commission mixte paritaire pour aboutir à un texte équilibré et pragmatique. Au delà de l’urgence, ce projet de loi contient déjà des réponses aux défis auxquels Mayotte Je tiens à saluer l’engagement de l’ensemble des parlementaires, ainsi que les apports précieux de ma collègue de groupe, Salama Ramia, actuellement à Mayotte, a relayé les attentes et les inquiétudes des Mahoraises et des Mahorais avec force et détermination. Ce projet de loi repose sur plusieurs piliers essentiels. d’abord la création d’un établissement public dédié à la reconstruction qui garantit une mobilisation forte de l’État tout en associant étroitement les élus locaux et les acteurs économiques de Mayotte. Il prévoit ensuite des assouplissements réglementaires pour pour accélérer la reconstruction, notamment des dérogations en matière d’urbanisme, d’accès aux matériaux et de commande publique en faveur des entreprises locales. Ces mesures visent à éviter les lourdeurs administratives qui pourraient freiner la relance tout en préservant un cadre rigoureux et transparent. Ce texte ne se limite toutefois pas aux infrastructures, il apporte un soutien direct aux Mahorais sinistrés par la suspension des cotisations sociales, la prolongation des droits aux allocations et des dispositifs fiscaux adaptés. Nous savons que la reconstruction ne peut se faire sans un accompagnement fort des familles et des entreprises durement touchées par la catastrophe. Je veux ici souligner le travail de solidarité et de dialogue qui a marqué cette commission mixte paritaire. Plusieurs points ont suscité des débats nourris, notamment l’implantation des locaux de services publics ou encore l’inscription des aides sociales et fiscales dans le temps. Ces échanges ont enrichi le texte et ont permis d’aboutir à des décisions équilibrées prenant en compte les réalités du terrain tout en évitant les écueils d’une approche purement dogmatique. Mayotte ne saurait pourtant être condamnée à l’urgence permanente : ce texte ne constitue qu’une première pierre

la régularisation foncière, l’accès à l’eau, l’éducation, au plus proche du quotidien de nos concitoyens mahorais. Mayotte n’a pas besoin d’une vision hors sol, il lui faut une politique ancrée dans ses réalités. La situation a atteint un point de saturation et nos décisions doivent être à la hauteur des défis. Mayotte n’est pas seule.

après les mesures d’urgence prises au lendemain du cyclone Chido, l’adoption de ce projet de loi est une nouvelle étape décisive et très attendue par Mayotte et ses habitants. Le groupe du RDSE votera, comme lors du scrutin précédent, les conclusions de la commission mixte paritaire. Tout au long de la discussion parlementaire, le Sénat s’est assuré que ce texte serait le plus possible élaboré à partir des besoins des Mahorais, et pour cause : la copie initiale du Gouvernement ne nous paraissait pas répondre pleinement à cette exigence. L’approche technocratique et verticale qui était privilégiée dans un texte rédigé à la hâte risquait de viser à côté de l’essentiel

La période de reconstruction qui s’ouvre doit aussi être l’occasion de repenser le dialogue entre la métropole et l’île. C’est en ce sens que la commission mixte paritaire a conservé dans son texte plusieurs mesures adoptées par le Sénat, afin que la reconstruction se fasse davantage en concertation J’ai ainsi à l’esprit l’article 1, qui renforce la représentation des collectivités locales dans la gouvernance du nouvel établissement public chargé de la reconstruction, la présidence est confiée par ailleurs au président du conseil départemental de Mayotte. La reconstruction de l’île prendra du temps, c’est certain, elle sera complexe, tant Mayotte accumule des difficultés structurelles depuis de nombreuses années : désordre foncier, pauvreté endémique, chômage élevé, pour n’en citer que quelques unes. Face à ce constat, le prolongement du dispositif relatif à la protection des entreprises et aux prestations sociales introduit par le Sénat est une réponse, certes temporaire, mais plébiscitée par les acteurs locaux. Sur la fiscalité, la discussion dans notre assemblée a permis d’introduire des dispositifs très attendus par les habitants, comme la création d’un prêt à taux zéro pour la reconstruction et l’extension de l’exonération de la taxe générale sur les activités polluantes à tous les déchets. Le texte issu de la commission mixte paritaire conserve l’équilibre trouvé au Sénat entre urgence et respect des libertés locales. Dans cet esprit, l’article 3, qui dispense d’autorisation d’urbanisme certaines constructions temporaires, a été réintroduit au Sénat dans une forme juridique plus sécurisée et son utilisation a été élargie aux écoles et aux bureaux administratifs.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, les débats que nous avons eus tout au long de l’examen de ce texte démontrent que la refondation de Mayotte doit reposer sur une discussion parlementaire exigeante. Le dialogue, l’écoute et l’association des acteurs mahorais sont les clés de réussite pour construire une voie de sortie apaisée pour l’île.